je vous remercie de votre invitation qui me permet de faire un point d'étape sur les discussions concernant notamment le plan de relance, ainsi que le prochain budget européen 2021-2027 et de répondre à vos questions à l'issue du débat.

Ce débat intervient à un moment très important- peut-être crucial -pour l'Europe et pour notre pays, car si l'épidémie n'a pas disparu, ses conséquences économiques et sociales apparaissent.

Plus personne ne remet en cause aujourd'hui le principe d'un plan de relance européen ambitieux. Chacun a également pris conscience que personne ne pouvait sortir seul de ce qui s'annonce comme la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si nous n'agissons pas vite et si nous n'agissons pas ensemble, nous irons vers une récession durable. Or nul ne peut se satisfaire d'une telle situation. Elle entraînerait l'aggravation des inégalités entre États et contribuerait à fragmenter le marché intérieur elle pourrait alimenter un déclassement économique durable de l'Europe et, surtout, elle pourrait mettre en péril des millions d'emplois et aggraver une situation sociale déjà difficile.

qui a été celle du Président de la République ces dernières semaines, car en diplomatie la méthode compte peut-être parfois plus que le contenu. contenu. La France et l'Allemagne ont proposé dès le 28 mai un outil de relance fondé sur la solidarité et sur un objectif bien compris et pleinement partagé de souveraineté européenne. Cet accord est l'aboutissement d'un très long travail de conviction mené par le Président de la République avec la Chancelière. Sans la main tendue par le Président à l'Allemagne depuis 2017, que ce soit au travers du discours de la Sorbonne, des rencontres à Meseberg, ou encore très récemment lors du conseil des ministres franco-allemand de Toulouse, nous n'aurions pas pu arriver à cette compréhension commune des moyens et de la nécessité de rendre l'Europe plus forte et plus souveraine. Je suis donc convaincue que s'il y a une victoire aujourd'hui, c'est celle de notre persévérance et de la persévérance du Président de la République à faire avancer le sujet d'une souveraineté européenne pleinement assumée et pleinement comprise au cours des dernières années. Suivant cette dynamique franco-allemande favorable, la Commission a proposé un cadre budgétaire complet le 27 mai. Nous pensons que cette proposition est à la hauteur de l'enjeu historique et qu'elle démontre une réelle ambition politique. Ursula von der Leyen a compris l'enjeu existentiel auquel l'Europe est confrontée. Notre responsabilité est maintenant de créer les conditions d'un accord dans les prochaines semaines en prenant en compte les besoins que chacun a exprimés. Ces besoins sont légitimes, car ils sont le reflet des situations politiques intérieures. Nous devons pleinement les apprécier.

C'est pourquoi nous multiplions les échanges avec nos partenaires. Le Président se trouve ce soir à La Haye pour un échange approfondi avec Mark Rutte. J'étais moi-même il y a dix jours en Autriche et, la semaine dernière, aux Pays-Bas. J'échange très régulièrement avec les pays du groupe de Visegrád et je me rendrai la semaine prochaine en Suède et dans les pays baltes.

Le premier concerne l'urgence. Nous avons une obligation de résultat pour les travailleurs, pour les entreprises. Ce plan de relance doit être opérationnel au 1 janvier 2021. S'il n'est pas prêt pour la relance, autant vous dire qu'il ne servira à rien.

Si nous réduisons la relance à un système de prêts, nous ne ferions qu'alourdir la charge pesant sur les pays les plus touchés et nous aggraverions davantage encore les distorsions au sein du marché intérieur. Je tiens à le dire très fortement il est question non pas de mutualiser les dettes du passé, mais d'investir ensemble dans les régions, dans les filières économiques les plus touchées, et cela au bénéfice de tous les États membres.

euro : c'est un critère essentiel pour créer de la convergence économique et de la synchronisation dans nos réformes plutôt que de la compétition. Nous devons à tout prix éviter de tomber dans un fonctionnement de type « troïka

sera essentiel. Nous souhaitons que ce plan de relance soit un plan condensé et non pas dilué. C'est pourquoi Bruno Le Maire a rappelé hier à Berlin que nous voulions que les fonds soient consommés en deux ans, en 2021 et en 2022.

Tous les acteurs devront se mobiliser, y compris les collectivités locales. Je sais votre connaissance fine des besoins de chacun de vos territoires. Il faudra nous pencher ensemble très rapidement sur la meilleure manière de nous assurer d'une consommation rapide des fonds mis à disposition. L'intérêt stratégique de la mission de simplification

Nous ne devons pas opposer reconstruire et investir. Le budget européen et le cadre financier pluriannuel, ou CFP, doivent être à la hauteur des ambitions de long terme. Je pense en particulier à des enveloppes qui contribuent à notre souveraineté, telles que celle de la politique agricole commune

réduire dans le temps le coût du remboursement de l'emprunt commun et mettre notre financement en cohérence avec nos objectifs, notamment environnementaux. C'est pourquoi nous demandons la fin

nous permettront d'investir ensemble sans augmenter le coût des contributions nationales. Pour conclure, je tiens à vous rassurer sur un point. Ce plan n'est pas fait en catimini.

européen aura aussi un rôle crucial à jouer dans l'élaboration du plan de relance national pour nos entreprises, nos territoires et nos citoyens. Vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui de l'ensemble des membres du Gouvernement pour conduire avec vous cette mission. Il me faut rapidement ajouter que la réunion de vendredi dernier a également permis aux chefs d'État et de gouvernement d'aborder la poursuite des négociations avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit, ainsi que le renouvellement des sanctions de l'Union européenne imposées à la Russie.

Madame la présidente, madame la secrétaire

En vérité, comme nous pouvions nous y attendre, le Conseil européen qui s'est tenu vendredi dernier n'a pas vraiment permis d'aboutir à un accord. Nous adhérons bien évidemment au au concept défendu par le Président de la République d'une Europe plus forte et plus souveraine, mais il y a encore loin des mots à la réalité. Vous avez décrit le risque d'absence d'un accord. Or le constat est terrible : une fois de plus, l'Europe a fait étalage de ses divisions, alors que les modalités de réponse à la crise sont en débat depuis mars dernier. Une décision rapide était pourtant absolument nécessaire. On évoque aujourd'hui un possible compromis en juillet, voire à la fin de l'été, mais vous l'avez dit vous-même, le temps presse. Après les annonces du mois dernier, 750 milliards d'euros serait allouée au plan de relance, la déception serait bien grande si les États se révélaient incapables d'aboutir. L'enjeu est économique, bien sûr, mais il est aussi politique, et il aura des conséquences sur la perception que nos concitoyens auront du rôle de l'Europe. La crédibilité de l'Europe est en cause. Si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord aujourd'hui face à une crise d'une telle ampleur, quand serons-nous véritablement capables de faire avancer l'Europe ? Y a-t-il eu des avancées lors de la réunion du Conseil de la part des pays dits « frugaux » ? Le Président de la République- vous l'avez dit -est en ce moment même aux Pays-Bas pour tenter de convaincre l'un de ces pays les plus réticents.

la relance. Quel contresens stratégique ! Nous avions pourtant la possibilité d'accompagner cette relance ô combien nécessaire. Où sont les 17 milliards d'euros qui étaient proposés il y a seulement deux ans par la Commission pour le Fonds européen de la défense et pour la mobilité militaire ?

Sous l'autorité de mon collègue Jean Bizet, je participe à un groupe de suivi qui entendra Michel Barnier jeudi prochain. Nous sommes très intéressés par cette audition, mais en vérité, nous sommes inquiets. Les négociations avec la Grande-Bretagne sont dans l'impasse.

le seul partenaire qui fixe à la défense les mêmes objectifs et lui alloue les mêmes moyens que notre pays. Le Sénat va s'y employer sur le plan parlementaire, car beaucoup de choses resteront à reconstruire avec le Royaume-Uni. Cette coopération doit rester au cours des prochaines années l'un des moteurs de la construction d'une défense européenne, à laquelle le Royaume-Uni a naturellement vocation à participer. Madame la secrétaire d'État, tout en rendant encore une fois hommage à votre détermination, comprenez que nous doutions de cette volonté d'aboutir de la part d'un certain nombre de nos partenaires, même si nous espérons encore. La parole

les États membres n'ont pas réussi à progresser ni sur la détermination du prochain cadre financier pluriannuel ni sur la mise en oeuvre d'un fonds de relance pour surmonter la crise actuelle. Cet ordre du jour ambitieux s'inscrit au coeur des compétences de la commission des finances. En effet, celle-ci a examiné la semaine dernière, sur mon rapport, une proposition de résolution européenne sur ce sujet, devenue hier résolution du Sénat, présentée par le président Jean Bizet et Simon Sutour, au nom de la commission des affaires européennes. Les débats au sein de la commission des finances ont souligné le caractère novateur de la proposition de la Commission européenne. Cette proposition, qui repose sur un couple formé par un CFP socle et un fonds de relance, présente deux avantages indéniables. Premièrement, elle permet d'augmenter significativement la puissance de feu du budget européen sans peser à court terme sur les contributions nationales. Deuxièmement, elle a le mérite de tenter de réconcilier plusieurs visions de cet attelage que constituent le CFP et le fonds de relance,

Toutefois, la commission des finances n'a pas donné de satisfecit tant les incertitudes et les points d'inquiétude demeurent nombreux. Le premier d'entre eux concerne le calendrier des négociations. Alors que le Conseil européen de la semaine dernière a surtout permis de constater des désaccords déjà bien connus, le temps presse pour mettre la prochaine programmation financière sur les rails. Les négociations se sont ouvertes en 2018, avec l'objectif d'éviter des retards importants pour la mise en oeuvre des programmes opérationnels en début de CFP tels que nous en avions connu en 2014. Madame la secrétaire d'État, un accord entre les États membres en juillet vous semble-t-il à portée de main ? Dans le cas inverse, quelles mesures seraient alors prises pour assurer la continuité du budget européen ? J'en viens au deuxième La Commission relève que l'articulation du budget européen augmenté du fonds de relance et des plans de relance nationaux est cruciale pour assurer la reprise économique. S'agissant des subventions prévues par la « facilité pour la reprise et la résilience », le calendrier de décaissement des crédits de paiement ne nous paraît pas adéquat. Le financement de la reprise doit intervenir dès le début du CFP. À cet égard, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous apporter des précisions- vous venez de le faire en partie -sur les projets d'investissement et les secteurs de notre économie qui pourront bénéficier en priorité du fonds de relance européen ? Notre commission s'est également inquiétée des modalités de remboursement de l'emprunt réalisé par la Commission européenne. À partir de 2028, deux pistes sont possibles : soit le remboursement est permis par la mise en oeuvre de nouvelles ressources propres de l'Union, soit il repose quasiment exclusivement sur une hausse significative des montants des contributions nationales des États membres. En la matière, rien n'est donc acquis. Or, en l'absence de certitude sur le remboursement dont devra s'acquitter la France, nous ne pouvons pas déterminer le taux de retour dont elle bénéficiera au titre du fonds de relance ni l'ampleur de la hausse à venir de sa participation au budget européen. La Commission européenne semble placer beaucoup d'espoir dans l'introduction d'un panier de nouvelles ressources propres. S'il est évident que cette solution offre une porte de sortie à un débat politiquement sensible, je crois qu'il est nécessaire d'aborder la question avec lucidité : malgré votre bonne volonté, l'Union européenne sera-t-elle en mesure de se doter de nouvelles ressources propres d'ici à 2028 eu égard aux réticences historiques des États membres en la matière ? portent notamment sur la proposition de création d'une ressource nouvelle reposant sur une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, ou encore sur celle de création d'une taxe sur le numérique. La Commission européenne a également proposé une taxe sur les grandes entreprises qui risquerait de peser sur le tissu économique européen. De plus, les recettes de plusieurs des ressources proposées ont vocation par nature à diminuer à mesure que les pratiques de consommation et de production évoluent, telles que les recettes de la taxe sur les déchets plastiques, ou encore les recettes issues de quotas d'émissions de carbone. La dernière inquiétude réside dans la progression du montant de notre contribution nationale à compter de 2021, et plus encore à compter de 2028. Dans un contexte de négociation marqué par le Brexit, les propositions initiales de la Commission européenne se seraient traduites par un ressaut de 6,9 milliards d'euros en moyenne par an. Cette hausse initiale n'incluant pas le remboursement du fonds de relance apparaît considérable compte tenu de la situation de nos finances publiques, encore plus dégradées à l'heure actuelle. Madame la secrétaire d'État, en cas d'impasse sur le volet des ressources propres, quelle sera la part de remboursement annuel du fonds de relance assumée par la France à compter de 2028 ? La

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen du 19 juin ouvre la voie à un tournant fondateur dans l'histoire de l'Union. Si aucun accord n'en a malheureusement expressément résulté, il n'a donné lieu à aucune remise en cause fondamentale de l'architecture générale de la proposition de la Commission européenne qui articule un projet révisé de cadre financier pluriannuel et un instrument de relance temporaire financé par un emprunt de la Commission, au nom de l'Union. Le premier serait doté de 1 100 milliards d'euros et le second de 750 milliards d'euros. Nous vivons ainsi un moment critique où se confrontent l'urgence de la crise entraînée par la pandémie de Covid-19 et le temps long de la construction européenne. Les Vingt-Sept s'accordent sur la nécessité d'apporter maintenant une réponse au choc économique provoqué par le confinement qui vient de prendre ou quasiment -, et c'est heureux. Or l'ampleur du choc et donc de la réponse à élaborer est telle qu'elle oblige à bousculer le cadre existant et conduit à échafauder un nouvel étage à l'édifice européen qui se construit dans la durée. La dénomination du nouvel instrument de relance telle que proposée par la Commission illustre ce paradoxe : c'est un plan de relance pour aujourd'hui, mais il se nomme « Union européenne de nouvelle génération car il engage l'Union sur trente ans. C'est en effet à cet horizon qu'est envisagé le remboursement de l'emprunt proposé. On conçoit donc l'extrême défi auquel étaient confrontés vendredi dernier les chefs d'État et de gouvernement encore réunis en visioconférence.

Sans doute ce moment n'est-il pas « hamiltonien » à proprement parler, puisqu'il n'est pas question que l'Union européenne reprenne les dettes des États membres dans un grand saut fédéral, mais il est certainement historique dans la mesure où les Ving-Sept envisagent de s'endetter ensemble pour le bien de l'Union. Ils reconnaissent ainsi leur attachement à la construction européenne et leur responsabilité commune envers l'avenir. C'est le fruit inattendu et « savoureux » de la crise profonde dans laquelle le virus a plongé notre continent. Il appartiendra ensuite aux Parlements nationaux, qui détiennent la souveraineté budgétaire, d'y consentir ou non. Avant d'en arriver là, beaucoup de sujets restent à régler. Car, au-delà de l'architecture globale du projet, l'essentiel est semble-t-il d'optimiser cet effort financier pour qu'il fortifie réellement l'Union européenne et lui garantisse une autonomie stratégique sur la scène mondiale. Concrètement, cela implique des arbitrages précis. Je pense d'abord à des arbitrages au service de la souveraineté alimentaire, qui repose sur nos agriculteurs. agriculteurs. Ces derniers ont besoin de garder le soutien qu'ils reçoivent du premier pilier de la politique agricole commune et d'être accompagnés dans les sauts technologiques contribuant au verdissement des pratiques agricoles. Ensuite, les arbitrages doivent servir la souveraineté industrielle, qui passe bien sûr par la relocalisation de chaînes de production stratégiques, comme en matière sanitaire, mais aussi par le déploiement des réseaux mobiles 5G dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et par une protection suffisante de nos entreprises stratégiques

ce qui suppose qu'il s'accompagne d'une modernisation de la politique de la concurrence, ainsi que d'une optimisation et d'une réactivité accrue de nos outils de défense commerciale. Je sais que c'est « en marche », si je puis dire.

J'aimerais bien que l'Union européenne se dote du même outil. Il reste aussi à s'accorder sur les modalités de mise en oeuvre du plan de relance. Certes, le principe d'un emprunt de la Commission au nom de tous semble acquis, mais les modalités de mise à disposition des États membres des fonds ainsi levés, par le biais de prêts ou de subventions, demeurent un sujet de discorde. Il en est de même des modalités de remboursement de cet emprunt, qui impliquent la création de ressources propres. Comment s'accorder sur un budget sans savoir comment il sera financé ? De ce point de vue, on peut comprendre la frilosité des États dits « frugaux », même si des considérations de politique intérieure expliquent en partie leurs postures, notamment en ce qui concerne les Pays-Bas.

l'épidémie de Covid-19 conduisant l'Europe, comme le reste du monde, au confinement de sa population affecte durement l'économie du continent : une récession attendue autour d'au moins 8,7 % pour la zone euro en 2020, une baisse des exportations de l'Union européenne estimée entre 9 % et 15 %, plusieurs millions d'emplois menacés. Selon les experts, nous serions face à la pire des crises connues en temps de paix. Aussi, nous sommes dans une situation d'urgence économique- c'est peu de le dire. Cette situation exige plus que jamais l'exercice concret de la solidarité entre pays, un principe théoriquement gravé dans le marbre. Doit-on en effet rappeler aux pays dits « frugaux » l'article 3 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que l'Europe « promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres » ? Certes, les propositions de la Commission européenne concernant l'instrument de relance sont ambitieuses et, à ce titre, on peut comprendre qu'elles suscitent des crispations. 750 milliards d'euros sous la forme de subventions et de prêts aux États membres les plus touchés par la crise sur le fondement d'un emprunt communautaire : osons le dire sans tabou, nous sommes sur la voie d'une dette européenne mutualisée. Le RDSE salue cette avancée qui nous semble indispensable pour garantir la cohésion de la zone euro. L'heure n'est plus aux tergiversations. Comme l'a rappelé la semaine dernière la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), « plus vite le paquet sera adopté, mieux ce sera pour l'économie de l'Union Même si l'on peut saluer l'esprit d'ouverture des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark et de l'Autriche, nous savons que la répartition entre subventions et prêts les préoccupe. Pourtant, c'est bien à l'aune du niveau des subventions que sera jugée la capacité de l'Europe à garantir enfin un véritable soutien mutuel entre États membres. Il faut donc s'en tenir à la proposition franco-allemande de 500 milliards d'euros sous la forme privilégiée de subventions. Déjà 540 milliards d'euros de prêts sont engagés au titre des premières mesures de soutien.

Si c'est le prix à payer pour obtenir un accord rapide et, surtout, le maintien d'un instrument reposant principalement sur des subventions, nous devrons nous y résoudre. Cette fameuse question des rabais me conduit à revenir sur le prochain cadre financier pluriannuel auquel est adossé l'instrument de relance. Les mêmes pays ont demandé une révision à la baisse de son montant global. Sur ce point, madame la secrétaire d'État, quelle marge de manoeuvre avons-nous ? La proposition de CFP du 27 mai est déjà assise sur un compromis. Raboter les 1 100 milliards d'euros sur la table ne permettrait pas de concilier les politiques traditionnelles et les nouvelles priorités. Il a déjà fallu consentir des sacrifices dans certains domaines par rapport à ce que l'on aurait pu faire avec la proposition de la Commission européenne de mai 2018, laquelle- je le rappelle -prévoyait une enveloppe de 1 279 milliards d'euros.

mais nous restons au-dessous du niveau du CFP en cours, alors que des filières agricoles, comme la viticulture ou l'horticulture, connaissent des difficultés considérables dans plusieurs États membres. Avec 8 milliards d'euros, le Fonds européen de la défense est également sacrifié sur l'autel des économies, dans un contexte stratégique pourtant très sensible. Par ailleurs, l'épidémie de Covid-19 impose une nouvelle priorité qu'il faudra doter de moyens : l'ébauche d'une Europe de la santé. Si l'organisation des systèmes de soins est une compétence exclusive des États, les traités ont toujours préconisé d'encourager un niveau élevé de protection de la santé des Européens. Nous voilà aujourd'hui face à cette nécessité. Je salue donc les efforts engagés en faveur du programme de l'Union européenne pour la santé dans le prochain soit 9,4 milliards d'euros au total. J'espère, en outre, que la politique européenne de la santé permettra de répondre à la question de la dépendance européenne à l'égard de l'Asie pour des biens aussi fondamentaux que le matériel médical et les médicaments. Le chantier est en tout cas ouvert ; on peut s'en réjouir. Tous ces engagements, avec pour toile de fond la transition verte, à laquelle mon groupe souscrit naturellement, supposent un réel effort financier dans la durée. S'agissant de l'instrument de relance, si le remboursement du capital n'intervenait qu'à partir de 2028 pour trente ans, il faudrait néanmoins envisager rapidement de nouvelles recettes pour ne pas alourdir les contributions nationales dans un contexte qui conjugue récession, départ du Royaume-Uni et probable maintien des rabais. Dans ces conditions, il faut aboutir rapidement à un accord sur un panier de nouvelles ressources propres. Lundi dernier, la commission des budgets du Parlement européen a une nouvelle fois demandé au Conseil de les mettre en oeuvre. Le dossier de la taxe sur le numérique semble faire son chemin. C'est une bonne chose, et mon groupe y est favorable, mais cette taxe ne rapporterait que 5 milliards tout comme la taxe sur les déchets plastiques. Un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'Union européenne est aussi attendu. Enfin, madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la question du filtrage des investissements. L'Europe s'apprête à déverser beaucoup d'argent pour sauver son économie, dont une majeure partie sera orientée vers les entreprises. Dans cette perspective, il est fondamental de mettre en place un instrument pour protéger les marchés européens. Le mécanisme de filtrage émergera-t-il avant la fin de l'année ? Mon groupe attend aussi beaucoup de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union face à la Chine, qui a été publiée en 2019, mais qui peine à se concrétiser, comme l'ont constaté les dirigeants européens réunis sur ce sujet le 22 juin dernier. Mes chers collègues, pour conclure, je rappellerai cette fameuse citation de Robert Schuman donnant le coup d'envoi à la Communauté européenne : « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. À l'aube de la plus grave crise économique qu'elle a connue, l'Union européenne a plus que jamais besoin d'unité et de solidarité. Mon groupe espère que tous les États membres seront au rendez-vous de ces deux principes fondateurs du pacte européen.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la vie en « distanciel » n'est pas la vie en « présentiel ». Et en politique, comme ailleurs, nous en faisons tous quotidiennement la délicate expérience. Difficile, en effet, de faire une campagne de proximité en distanciel à l'occasion du second tour des élections municipales, qui aura lieu ce dimanche. Difficile également de mener une réunion de commission tant soit peu dynamique, de garder toute son attention lors de marathons virtuels, qui nous conduisent parfois à participer à quatre ou cinq téléconférences dans la même journée. En dehors des interférences dues à certains micros que l'on oublie de couper, finis la spontanéité des échanges, les petites pauses et les apartés informels, deux à deux, qui permettent souvent d'esquisser un début de compromis ou de rapprochement. mot « distanciel »- cela ne vous aura pas échappé -, il y a le terme « distance ». Et s'il est vrai que la communication en distanciel permet bel et bien aux différents points de vue de s'exprimer, ce « cadre particulier de l'expérience », pour reprendre une expression chère au sociologue Erving Goffman, ne permet guère en revanche de construire une relation véritablement interactionnelle et authentiquement dialogique. Que signifie, en effet, un silence dans un échange distanciel et médiatisé par les nouvelles technologies de l'information ? Approbation, désapprobation, réflexion, inattention ou, tout simplement, problème de transmission ou de réception ? Cette délicate expérience du distanciel est celle que les vingt-sept chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les principaux dirigeants de l'Union ont pu vivre à l'occasion du sommet virtuel qui s'est tenu vendredi dernier. Mais cessons de geindre et de laisser croire que les maigres résultats qui ont résulté de cette réunion seraient le seul fait de la technologie employée. Certes, la délicate question du prochain cadre financier pluriannuel et du plan de relance européen aurait peut-être pu connaître quelques avancées supplémentaires si ce Conseil avait eu lieu en présentiel. Mais rappelons quand même que les discussions autour du cadre budgétaire 2021-2027 durent depuis plus de deux ans et que, pour l'essentiel, elles se sont déroulées en présentiel, sans que le résultat final soit aujourd'hui clair, et ce à six mois à peine de la mise en oeuvre effective

de paquet budgétaire qui n'a- il faut le souligner -qu'un tout petit mois d'existence. En dépit de cet étrange sommet « pour voir », il faut dire aussi que nos diplomaties respectives n'ont, en amont et en aval de celui-ci, pas chômé pour faire avancer les positions des uns et des autres. Parties à deux le 18 mai dernier, la France et l'Allemagne ont vite été appuyées par la Commission et suivies par une large majorité des États membres. Dans ces délais inaccoutumés à l'échelon de l'Europe, c'est déjà en soi un petit miracle Par ailleurs, et même s'ils formulent certaines réserves, c'est sans doute la première fois depuis plusieurs années que les pays du groupe dit de Visegrád ne sont pas au coeur de l'opposition à un procès d'approfondissement et de renforcement de l'Union européenne. Bel exploit ! ! Autre point positif, c'est l'Allemagne- elle prendra la présidence du Conseil le 1juillet prochain - qui sera à la manoeuvre lors des négociations finales sur ce grand paquet budgétaire.

Ceux qui connaissent bien l'histoire de la construction européenne savent que les accords européens les plus importants ont toujours été conclus, par le passé, sous les auspices de la présidence d'un des grands pays membres de l'Union. Au-delà des belles raisons d'espérer que je viens d'énoncer, on ne peut cependant pas occulter les actuels points de tension qui se font jour entre États membres, au premier rang desquels figurent les fortes réticences exprimées par les fameux pays dits « frugaux Peu ou prou, ces derniers contestent le recours à l'emprunt européen pour financer ce plan ou, tout au moins, la répartition entre subventions et prêts, qui penche actuellement nettement en faveur des premières. Bénéficiaires de rabais sur leurs contributions nationales, ils refusent leur suppression en dépit du départ du Royaume-Uni. Ils insistent sur l'instauration de conditions pour les pays qui devraient principalement bénéficier de ce plan de relance : un semestre européen plus exigeant et l'engagement d'importantes réformes structurelles par les pays bénéficiaires. La question des ressources propres est centrale et même la clé de voûte d'un accord. Sans nouvelles ressources propres, le remboursement de la dette européenne risque, à terme, d'échoir principalement aux pays contributeurs nets au budget de l'Union. Et comme les décisions concernant les ressources sont adoptées tous les sept ans, à la fin de chaque cadre financier pluriannuel, un changement en profondeur dans ce domaine doit, selon les règles européennes, passer par la procédure législative spéciale, qui requiert l'unanimité du Conseil, la ratification du Parlement européen et celle des parlements nationaux. Au sein du club des quatre « frugaux », les positions ne sont heureusement pas toutes aussi fermes qu'il y paraît à première vue. La Suède et le Danemark pourraient être plus conciliants que l'Autriche et, surtout, les Pays-Bas. Concernant l'Autriche,

Le cas des Pays-Bas est plus délicat, car l'euroscepticisme est puissant dans l'opinion. Le Premier ministre, Mark Rutte, est actuellement à la tête d'une coalition assez hétérogène, qui ne dispose que d'un siège de majorité à la seconde chambre des États généraux. Pour autant, les nouvelles du jour semblent laisser quelques espérances, si j'en crois un article paru cet après-midi dans un grand quotidien du soir. Le déplacement du Président de la République ce soir à La Haye pour rencontrer Mark Rutte n'est sans doute pas étranger à cette soudaine évolution. Bien sûr, et comme toujours dans une négociation européenne, il y aura certainement des concessions réciproques pour parvenir à un accord. Madame la secrétaire vous êtes indubitablement combative, mais êtes-vous indubitablement optimiste quant à l'obtention d'un accord au sein du Conseil européen avant la fin du mois prochain ? Plus précisément, quelles sont les concessions acceptables qui vous semblent pouvoir être faites pour y arriver ? La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen était chargé d'adopter d'un même mouvement la nouvelle proposition de cadre financier pluriannuel et le plan de relance annoncé par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Ses résultats sont loin de correspondre aux élans d'enthousiasme vus ici ou là pour saluer l'étape historique que serait en train de franchir l'Union européenne face à la crise du Covid-19. Certes, l'ampleur de la crise oblige les États membres, le Conseil et la Banque centrale européenne à réagir de manière inédite, faisant d'ailleurs voler en éclats des tabous budgétaires et monétaires qu'on nous disait indépassables il y a quelques mois encore. Mais empêtrée dans son modèle compétitif et concurrentiel, arcboutée contre l'augmentation des dépenses sociales et publiques, sans lesquelles pourtant le désastre sanitaire aurait été plus grave encore, l'Union européenne affiche toujours les mêmes divisions, les mêmes concurrences et, surtout, la même incapacité à se projeter résolument dans un nouveau modèle solidaire, tourné vers l'avenir, le développement de la sécurité humaine et de la protection de la planète. Un constat s'impose : aucun accord définitif n'a été trouvé au Conseil européen. On entre manifestement dans un marathon de négociations qui va durer tout l'été, et dont il faudra suivre les compromis successifs pour se faire une idée finale. Première remarque : l'addition du CFP et du plan de relance masque les évolutions structurelles du cadre financier pluriannuel, globalement en recul, au détriment notamment de la PAC et des fonds de cohésion. On nous explique que le plan de relance fait davantage que compenser. Mais le maquis de l'accès aux nouvelles lignes budgétaires va encore se compliquer- et non se simplifier, madame la secrétaire d'État ! -, et les destinataires ne seront plus forcément les mêmes. Les inquiétudes persistent donc.

joué un rôle important pour imposer aux États membres les politiques d'austérité si durement payées pendant la crise. Je pense notamment aux systèmes de santé publique ou au secteur de la recherche.

Aurons-nous un vrai débat, transparent, sur la gestion de ces fonds ou nous imposera-t-on une répartition dictée par les mécanismes budgétaires européens d'avant-crise ? Par exemple, pour la santé et la recherche, qui devraient être des priorités absolues après ce que nous venons de vivre, les sommes restent modestes : le fonds Santé est doté de 9,4 milliards d'euros pour toute l'Union européenne, alors que les besoins excèdent cette somme sur la période pour notre seul pays. La France ne doit-elle pas tenter de flécher avec plus de rigueur cet argent, afin de financer prioritairement le développement d'investissements publics dans la transition écologique des secteurs de l'énergie, des transports, notamment ferroviaires,

Présenté comme une solution européenne aux défis de la 5G, voilà un groupe auquel nous avons vendu Alcatel, qui est gavé depuis des années de subventions publiques et d'exonérations fiscales et sociales, et qui annonce la suppression de plus de 1 000 emplois dans le secteur de la

il faut revoir en profondeur tous les critères pour en finir avec un système de conditionnalité draconien pour les dépenses sociales et publiques et d'inconditionnalité pour les grands groupes, qui mangent aux deux râteliers : les subventions publiques, d'un côté, le dumping social et l'évasion fiscale, de l'autre. Pour réussir la relance, il ne suffira pas de brandir des chiffres, aussi nécessaires soient-ils. L'enjeu est de savoir quel sera le modèle sur lequel s'appuiera le fonds de relance : le modèle compétitif du monde d'avant

C'est une véritable victoire pour nos peuples et notre destin commun. Nous venons de faire un pas important en faisant le choix de sortir vite et ensemble de cette crise. Nous ne pouvons que nous en réjouir et être fiers de nos accomplissements que l'histoire, j'en suis sûre, jugera à la hauteur de ce que nous venons de réaliser. Faire le choix de mutualiser notre dette, financée en partie par des ressources propres, bien construites, vertes, sociales et rétablissant l'équilibre recherché. Se mettre d'accord sur un budget européen puissant, donnant à l'Union les moyens de ses ambitions est un signe que cet espoir européen si nécessaire Les politiques historiques, tout comme les nouvelles priorités, seront financées de manière équilibrée. « Ensemble, elles permettront aux citoyens européens d'avoir accès à une alimentation de qualité, de développer des projets dans nos territoires, de créer et de produire ensemble dans un tissu industriel innovant, d'agir pour notre protection commune, d'avoir accès à un numérique sain et encadré et, enfin, de vivre dans une Europe où l'impact sur la planète est mesuré, permettant aux générations futures d'entrevoir un avenir, qu'il y a quelque temps encore elles pensaient si sombre. L'Europe tient finalement le rôle de phare qu'elle se dessine depuis de nombreuses années. Enfin, nos relations futures avec les Britanniques seront claires et apaisées pour que nous contribuions ensemble à la progression du continent européen, à la construction et au respect de nos valeurs communes. » Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme j'aurais aimé pouvoir tenir ce discours ce soir Bien sûr, nous savions tous qu'il n'y aurait pas d'accord vendredi dernier. Le Conseil européen nous laisse tout de même espérer une issue favorable, tout en nous mettant en garde sur les difficultés qu'il reste à surmonter. Mais n'est-ce pas la définition même de l'Europe ? Ce soir, cependant, l'Européenne convaincue que je suis souhaite tout de même murmurer ce rêve d'Europe, ce rêve qui est à réaliser demain. Demain, c'est désormais le sommet de la mi-juillet.

Je suis également en faveur de ressources propres, issues notamment d'une taxation du numérique, du plastique et du carbone, afin de financer cette relance, mais aussi le budget pluriannuel. Concernant ce budget, nous sommes toujours en faveur d'un budget fort et équilibré entre les nouvelles orientations politiques de la Commission européenne et les politiques historiques : les unes ne peuvent aller sans les autres et la réciproque est vraie.

de subventions, de répartition, d'ampleur du budget, ou encore de maintien des rabais, pour ne citer que ces sujets, et, je veux le dire, ces interrogations sont légitimes. Nous comprenons les volontés, les enthousiasmes, les peurs, les résistances ... et les calendriers aussi

nous avons besoin d'une Europe forte. Nous devons retrouver une Europe sereine, juste et prospère, pour que les Européens, en plus de tirer fierté de leur modèle, puissent continuer à créer et vivre ensemble. Je connais votre engagement européen, madame la secrétaire d'État, ainsi que celui du Gouvernement. C'est pourquoi je ne peux que vous assurer, ce soir, de notre soutien dans les négociations qui se profilent et souhaiter une réussite européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, pourrait proposer un plan de relance amendé lors de la prochaine rencontre, prévue dans le courant du mois de juillet. Quelles sont les lignes rouges pour la France ? Les représentants des Pays-Bas et de la Suède ont déjà affirmé qu'un accord avant la pause estivale n'était ni probable ni forcément souhaitable. Quelle est la position de la France, compte tenu de la longueur du processus décisionnel en Europe, notamment de la nécessité de ratification par les États membres ?

Je souhaite saluer le travail considérable du négociateur européen en chef, Michel Barnier, et de ses équipes. Là encore, un accord n'est pas envisageable. Un, que nous voyons de nouveau se profiler, ne l'est pas davantage, même si nous devons nous préparer à cette éventualité. Le dossier du secteur de la pêche est important, tout comme l'est la nécessité d'un accord global et de règles justes et équilibrées de libre concurrence entre les deux acteurs. La situation des citoyens européens et britanniques l'est tout autant, comme celle des entreprises. Mais ne soyons pas naïfs non plus ! Nous devons faire de cette séparation un levier de coopération et de lutte conjointe pour la préservation de nos valeurs communes. Le Royaume-Uni reste notre allié et notre ami. Faisons en sorte que notre future relation repose sur des bases claires et nous permette de tisser de nouveaux liens dans le respect, à la fois, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Madame la secrétaire

Certes, mais cela était attendu, le Conseil n'a pas abouti à un accord sur le plan de relance. Cependant, cette rencontre a montré que le dialogue est possible, malgré les différentes lignes de fracture traversant le continent. Le maintien d'un dialogue constructif entre les dirigeants des Vingt-Sept est bien sûr essentiel sur le fond, mais également crucial sur la forme. En effet, comme l'a rappelé le Président de la République, il serait dangereux de présenter à nos opinions publiques l'image d'une Union en proie aux conflits ouverts, alors que l'Europe traverse des heures sombres et que les citoyens exigent des mesures fortes, rapides et claires. Parmi les fractures européennes, la plus nette en l'espèce est évidemment celle qui partage l'Union européenne entre le Nord et le Sud. Depuis plusieurs mois, nous voyons que les pays du Nord, pays « frugaux » en tête, campent sur leur position, en défendant un cadre financier pluriannuel limité à 1 % du PIB de l'Union et la nécessité de coupler les aides économiques à des réformes structurelles. En face, ceux du Sud, en particulier l'Italie et la France, plaident pour une véritable solidarité européenne, qui bénéficierait à l'ensemble du continent. Le fait que Berlin s'entende avec Paris pour défendre une position alignée sur les souhaits de Rome, ou encore de Madrid, est en soi un événement. Il permet, en outre, de faire véritablement bouger les lignes entre Européens, ouvrant la voie à un accord. Pour l'Alsacien et l'Européen que je suis, retrouver un couple franco-allemand ambitieux et force de proposition ne peut que constituer une excellente nouvelle, surtout après ce que nous avons vécu pendant le confinement

Le cadre financier pluriannuel en discussion doit être adapté pour permettre à l'Union européenne de faire face aux conséquences de la crise que nous traversons. Nous espérons donc que l'accord sera conclu rapidement, dans l'intérêt de nos entreprises et de nos territoires.

Les agriculteurs ont fait la preuve de leur résilience durant la crise et surtout, s'il en était besoin, de leur rôle absolument essentiel pour notre société. Si l'Europe n'a pas connu de pénurie, malgré le confinement pratiquement généralisé du continent, c'est grâce à eux ! Je souhaite, à ce titre, les saluer. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Doter l'Europe des moyens de sortir de cette crise plus forte qu'elle n'y est entrée : voilà l'enjeu des discussions qui doivent se poursuivre cet été

Même si nous considérons que le plan de relance reste en deçà de la gravité de la crise et des menaces pesant sur l'économie européenne, il n'empêche qu'il innove, dans sa conception comme dans ses modalités.

Ce plan a donc le mérite de marquer un pas qualitatif dans l'approche budgétaire européenne. Pour nous, il a deux vertus.

que toutes les crises ont fait avancer l'Europe. Si, aujourd'hui, nous disposons d'une politique régionale et de fonds structurels, nous le devons aux Britanniques, qui avaient marchandé, au début des années 1970, l'acceptation de la

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire a pris l'Europe de court. Sur un continent déjà en proie au doute, après l'effondrement de la Grèce, la crise migratoire, la vague de terrorisme, le Brexit,

du « malade européen » au prix d'un endettement lourd. Cette pandémie, c'est d'abord, je crois, la fin d'une illusion. L'Union européenne n'est pas une bulle prospère, protégée du monde par la seule vertu du droit et des valeurs. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Elle est interdépendante, au contact d'un monde en crise et en compétition. Ce n'est pas un monde de « Bisounours », pour reprendre le terme récent d'Hubert Védrine. La question de la sécurité des frontières reste primordiale. Les Européens ne devront plus tergiverser pour les fermer en cas de besoin. À ce titre, la reprise de l'épidémie en Chine appelle à la prudence. Soyons réalistes et mesurons l'accroissement des risques sanitaires, environnementaux ou géopolitiques La probabilité de récurrence d'événements graves devrait s'accroître et aujourd'hui, à tort ou à raison, là aussi, aucun citoyen ne répond spontanément que l'Europe protège. Or, dans le monde de demain, il faudra peser. Même si on peut le déplorer, il nous faut intégrer le durcissement des relations internationales, qu'elles soient politiques ou économiques, y compris dans nos rapports avec certains de nos alliés extracommunautaires et, en retour, très probablement, durcir notre posture. La relance massive de l'économie européenne ne servira à rien si elle ne s'accompagne pas d'un changement d'état d'esprit. Partout ailleurs, lorsque les intérêts sont menacés, les États n'hésitent pas à préserver leurs filières et leurs entreprises : préférences, mesures douanières, extraterritorialité du droit, etc. Dans ce contexte, l'Union européenne continue à présenter l'ouverture de son marché sous un seul jour bénéfique. Pourtant, le partenariat transatlantique, le Mercosur, les accords avec le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ont fini par susciter de vives inquiétudes, notamment en France, tant des consommateurs que des filières agricoles. L'Union européenne poursuit néanmoins sur cette voie, avec un accord commercial avec le Mexique, au moment où chacun aurait pu penser que la crise sanitaire amènerait à envisager la mondialisation autrement. Dans les domaines sanitaire ou militaire, notamment, l'approbation par la France de l'axe franco-allemand ne doit pas emporter pour seule conséquence le renforcement des groupes industriels allemands. Il faut créer les conditions en France d'une réindustrialisation et mieux protéger les entreprises des prédations étrangères, en particulier extraeuropéennes, afin que le concept d'autonomie stratégique ne reste pas un vain mot. Sur le plan environnemental, l'engagement de l'Union européenne en faveur du climat et des énergies renouvelables ne doit pas conduire à s'enfermer dans un choix entre les éoliennes chinoises ou allemandes. Les actions en vue d'améliorer la résilience des systèmes de santé, d'accroître la promotion de l'innovation dans le secteur de la santé en Europe sont bienvenues, mais pourront-elles faire pièce aux moyens considérables des routes de la soie de la santé chinoises et limiter notre dépendance à la Chine pour certaines molécules ou certains équipements sanitaires ? La somme des événements récents doit aussi amener un tournant pour l'Europe de la défense. Aux États-Unis, l'industrie de défense ne s'est pas arrêtée pendant l'épidémie et elle bénéficie d'un plan colossal de soutien, quand le budget du Fonds européen de la défense donne lieu, lui, à d'inquiétants atermoiements. En réalité, il sert de variable d'ajustement

Compte tenu, d'une part, de la réaffirmation des grandes puissances et des acteurs régionaux, d'autre part, du montant des dettes engagées pour surmonter la crise sanitaire en Europe, la secrétaire d'État, nous payer le luxe d'échouer. Ce serait à la fois déplorable et dangereux. L'Europe, c'est vrai, n'est pas parfaite elle doit être adaptée à ces nouveaux paradigmes. C'est, je crois, non pas aux hauts fonctionnaires européens de le faire, mais bien aux États qui la composent d'en être les moteurs. Si cette crise doit amener un progrès, c'est peut-être celui-là

été qualifié de première étape importante par certains, d'échec par d'autres. Une fois encore, la vérité se trouve sans doute entre les deux positions. ce sommet entérine un changement de lignes sur notre continent. Tout d'abord, il témoigne du retour d'un couple franco-allemand à l'initiative, donnant une impulsion politique politique nécessaire face à la menace existentielle de lignes de fracture irréconciliables qui s'étaient esquissées, en mars, entre le nord et le sud de l'Europe. Ensuite, si le plan de relance, post-crise sanitaire, mais pré-crise économique, a été discuté pour la première fois et s'il est encore loin de faire l'unanimité, il marque un tournant majeur dans l'intégration du continent : celui de l'emprunt commun. Face à une crise imputable à personne, mais affectant tout le monde, la logique d'une dette mutualisée permet de casser la logique de blocs qui empoisonne les discussions européennes, tout en traduisant une souveraineté commune, sur laquelle je reviendrai. S'agissant du cadre financier pluriannuel, je partage pleinement la position du Parlement européen : de nouvelles ressources fiscales propres à l'Union européenne permettant d'alléger les contributions des États membres sont indispensables. Plusieurs pistes sont à l'étude, et ce depuis de nombreuses années déjà. Il reviendra aux chefs d'État de trancher afin d'avancer. Je défends, pour ma part, la position, adoptée par le Sénat le 14 janvier dernier, d'une taxe carbone aux frontières, mais je suis également favorable à un élargissement des recettes collectées sur le marché du carbone européen, ou encore à une taxe sur les transactions financières, mesure également défendue par le Sénat depuis 2013. Madame la secrétaire d'État, concernant ce cadre financier et face aux nombreux sujets de désaccord, le maintien des rabais sera-t-il une des solutions pour, finalement, aboutir à un accord avant la fin de l'année ? Enfin, plus généralement, face à la crise sanitaire, l'Union européenne a choisi de se mettre en retrait, qu'il s'agisse de la suspension des règles budgétaires et du droit de la concurrence, du rétablissement des frontières, ou encore de la suspension des principales libertés Les États-nations ont dès lors recouvré leur souveraineté pour répondre à l'urgence de la crise. Mais face à la crise économique, il nous faut désormais investir à l'échelon européen une souveraineté nouvelle nouvelle : commerciale, en filtrant les investissements dans les secteurs stratégiques ; industrielle, en développant des projets importants d'intérêt européen commun ; stratégique, en s'affirmant comme un pôle d'équilibre entre les États-Unis et la Chine.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les chefs d'État et de gouvernement européens étaient réunis ce vendredi pour discuter du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, censé aider le vieux continent à sortir d'une récession historique. Comme il fallait s'y attendre, ce Conseil européen a une nouvelle fois mis au jour les profondes divergences entre les Vingt-Sept sur ce sujet. Les discussions achoppent toujours sur les modalités concrètes d'application de ce plan, que ce soit son volume total, la répartition des sommes, ou encore la nature des aides. Les discussions n'ont pas non plus beaucoup progressé concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période couvrant les années 2021 à 2027. Quand les pays dits « frugaux » souhaitent une baisse importante du budget des politiques traditionnelles et s'accrochent à leurs rabais, les autres pays, dits « amis de la cohésion », plaident au contraire pour un budget ambitieux et doté de ressources propres pour éviter les coupes envisagées dans le budget de la cohésion et de la politique agricole commune. À propos de cette dernière, saluons la majoration de 4 milliards d'euros sur le premier pilier et de 5 milliards d'euros sur le second, auxquels devrait s'ajouter un abondement de 15 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Cet effort sera toutefois loin de compenser la baisse de 8 % à 10 % du budget de la politique agricole commune en euros constants. Les Européens ne semblent toujours pas avoir pris conscience de l'importance stratégique de leur agriculture, alors même que celle-ci a démontré toute sa capacité à assurer l'approvisionnement alimentaire de 500 millions de consommateurs au plus fort de la crise ! À l'heure où l'on parle de relocalisation et de souveraineté retrouvée, n'oublions pas que le secteur agricole est l'un des rares domaines dans lesquels notre pays a gardé une réelle capacité à produire N'affaiblissons pas notre souveraineté alimentaire par des décisions hasardeuses, comme la proposition incompréhensible de la Commission européenne de baisser de 10 % la superficie des terres cultivables en Europe et, donc, en France. Pour revenir à l'instrument de relance au centre des discussions des Vingt-Sept, plusieurs propositions doivent être saluées, comme la création d'un nouveau programme de santé,, doté de 7,5 milliards d'euros et destiné à renforcer la sécurité sanitaire et à anticiper les futures crises. La concentration des engagements de dépenses sur une période courte- 2021-2024 -est également un choix bienvenu ; elle soulève néanmoins des enjeux importants en termes de capacité de mise en oeuvre, d'ingénierie et d'absorption des fonds. Ne reproduisons pas la technicité de la politique de cohésion, qui aboutit souvent à une sous-consommation des fonds européens. Enfin, la question des ressources propres de l'Union est un sujet majeur. La Commission souhaite les développer pour soulager les budgets nationaux et rendre le budget européen moins dépendant des contributions des États membres. Mais elle doit encore clarifier ses propositions et, surtout, veiller à maîtriser l'imposition globale pesant sur les ménages et les entreprises. N'ajoutons pas encore à l'overdose fiscale qui touche beaucoup de pays européens, à commencer par la France. L'Europe doit s'atteler rapidement au projet de barrière écologique aux frontières de l'Union européenne, comme l'a réclamé le Sénat dans une récente résolution soutenue par nos collègues Jean-François Husson et Bruno Retailleau. En taxant les produits provenant de pays qui s'affranchissent de toute réglementation environnementale, nous renforcerons la compétitivité de nos entreprises et de nos agriculteurs, soumis à des normes beaucoup plus exigeantes que leurs partenaires commerciaux. Pour conclure, mes chers collègues, je veux dire que les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront en juillet pour tenter de débloquer la situation. Il y a urgence, et vous l'avez dit, madame la secrétaire d'État. Un échec des négociations serait désastreux politiquement, il alimenterait les tendances nationalistes ; économiquement, il aggraverait encore la récession et la hausse du chômage. Les Européens sont donc condamnés à réussir, sous peine de discréditer définitivement le projet européen. Car l'Europe traverse depuis dix ans une succession de crises qui ont montré ses fragilités et ont accru la défiance des opinions publiques envers la construction européenne : crise économique et financière, crise sécuritaire avec la résurgence des attentats terroristes, crise migratoire, crise sanitaire. Nos pays étant interdépendants, chacun doit prendre conscience que la bonne santé économique de tous est dans l'intérêt de chacun ! Le prochain Conseil européen de juillet devra donc incarner cette indispensable solidarité européenne et montrer à nos concitoyens que l'Europe est capable de les protéger, enfin. Pour cela, elle doit réussir à dépasser ses divisions pour se hisser à la hauteur des enjeux auxquels notre continent doit aujourd'hui faire face. La parole est à M. Cyril Pellevat.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà près de soixante-dix ans que l'intégration européenne se poursuit et que les divers pays du continent européen collaborent, coopèrent et créent des liens toujours plus étroits. La construction européenne n'a cependant pas toujours été aisée et a connu son lot de complications. L'Union a traversé plusieurs crises, et nous ressentons encore aujourd'hui les effets de certaines d'entre elles. Mais, même s'il n'a pas toujours été facile de trouver des solutions satisfaisantes pour tous, l'Union européenne a jusqu'à présent réussi à les dépasser. Avec l'arrivée de la pandémie sur le territoire européen, nous sommes de nouveau confrontés à une crise majeure, risquant d'ébranler le modèle européen. Et si nous voulons nous en relever, une réponse forte et coordonnée est nécessaire. Cette collaboration a permis de faire aujourd'hui de l'Union européenne la deuxième puissance économique mondiale, et il faut tout mettre en oeuvre pour la maintenir à ce niveau, pour le bien de l'Union comme de la France. Mais si l'économie est une part essentielle de sa construction, l'Union européenne représente aussi le partage de valeurs et de principes démocratiques, d'entraide et de solidarité. Le respect de ces valeurs sera essentiel pour maintenir ce qui a été construit jusqu'à Il n'est pas possible, au regard de l'ampleur de la crise, de s'en sortir sans pouvoir compter sur nos partenaires européens, mais également sans qu'ils puissent compter sur notre soutien. Ainsi, la proposition de la Commission européenne d'adosser au cadre financier pluriannuel un instrument de relance, outil de redistribution et de solidarité, composé de 500 milliards d'euros de subventions et de garanties qui ne devront pas être remboursés, ainsi que de 250 milliards d'euros distribués sous forme de prêts, est une solution forte et satisfaisante, qui reflète ces principes sur lesquels l'Union européenne s'est bâtie. Des divergences entre les États membres se font pourtant sentir, et pour certains, dits « frugaux », l'absence de remboursement n'est pas envisageable. Ils estiment l'émission de prêts plus adaptée ou souhaitent voir ces subventions assorties de conditions, tel que cela avait été mis en place pour les pays en difficulté lors de la crise des dettes souveraines. Émettre uniquement des prêts ne me semble cependant pas envisageable, comme vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État. Assortir la distribution des subventions de conditions relatives au respect des priorités de la Commission- numérique, écologie, amélioration de la compétitivité économique -rappelle cependant de mauvais souvenirs aux pays ayant dû par le passé se plier à de nombreuses exigences, afin d'obtenir des prêts. En outre, la facilité pour la reprise et la résilience s'intégrera dans le cadre du semestre européen, ce qui impliquera en tout état de cause un dialogue exigeant entre les États membres et l'Union. Nous le savons, aucune proposition ne pourra pleinement satisfaire tous les États membres. Mais il est urgent de trouver une solution si nous souhaitons conserver la confiance des marchés financiers et éviter d'attiser un rejet massif du modèle européen par nos concitoyens, doutant de l'efficacité de l'Union. Par ailleurs, il est important de rappeler que les États-Unis prévoient un plan de relance trois fois plus important que le nôtre. Si nous ne parvenons pas rapidement à un accord, de grands groupes américains pourraient alors en profiter pour acquérir de larges parts de marché en Europe. Il devient donc de plus en plus impératif de trouver un compromis. Mais il faut aussi apprendre des erreurs du passé, et ne pas les reproduire. Ainsi, des conditions trop strictes ne me semblent pas envisageables. Il serait toutefois intéressant, afin de parvenir le plus rapidement possible à un accord, de consentir à poser certaines conditions, sans qu'elles soient trop lourdes pour les États, comme cela a pu être le cas par le passé. Ainsi, madame la secrétaire d'État, j'aurais aimé connaître votre position au sujet de cette conditionnalité des subventions.

bénéficieront ainsi d'un financement à hauteur de 205 millions d'euros. C'est un pas important, et l'on peut s'en réjouir. Pourtant, dans les discussions sur le cadre financier pluriannuel, le Fonds européen de la défense apparaît toujours comme une variable d'ajustement. En février dernier, Gisèle Jourda et moi-même avions présenté une proposition de résolution européenne qui soulignait la nécessité, si l'on veut réellement assurer l'autonomie stratégique de l'Union et renforcer sa base industrielle et technologique de défense, de doter ce fonds à la hauteur initialement prévue.

faisant oublier son intransigeance dans la crise financière grecque- c'était il y a seulement cinq ans. Aujourd'hui, elle s'emploie à convaincre les États d'Europe du Nord d'accepter la création d'un nouvel instrument de relance.

la légalité de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne, menaçant ainsi la survie de l'euro. Dans dix jours, l'Allemagne prendra la présidence du Conseil de l'Union.

l'Allemagne dépend de celle de ses clients et de ses fournisseurs. Cela étant, on ne peut manquer de s'inquiéter de la pérennité de l'engagement européen de notre plus proche voisin, au regard des tensions qu'il provoque, et dont le tribunal constitutionnel de Karlsruhe donne un puissant écho.

La rencontre, la semaine dernière, entre Boris Johnson et les présidents du Conseil européen et de la Commission n'a pas porté les fruits espérés. Londres refuse d'étendre la période de transition : dont acte. Les pourparlers avec les Britanniques butent encore et toujours sur ces quatre sujets : les conditions d'une concurrence équitable- le fameux -, l'accès de nos pêcheurs aux eaux britanniques, la gouvernance future de l'accord et la coopération judiciaire et policière.